que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes ; l’orateur disposera alors à son tour d’un droit de réplique, pour une minute.

Vous le savez sans doute, une proposition de loi visant à reconnaître le bénévolat de sécurité civile a été déposée à l’Assemblée nationale en avril 2023, avant d’être adoptée à l’unanimité par la commission des lois, puis en séance publique en mars 2024. Elle était défendue par le député Yannick Chenevard, qui est présent ce soir dans

Vous incarnez toutes et tous le visage d’une France solidaire, ouverte, généreuse, […] et je suis fier de cette énergie que chacun de vous déploie en ces moments difficiles et éprouvants, par le seul souci de l’autre et le seul intérêt de la France.

Ils agissent dans un cadre préventif, par exemple en assurant le secours lors de manifestations ou événements, mais aussi en dispensant des formations et en conduisant des actions de sensibilisation aux risques et aux réflexes de premiers secours.

Le texte adopté à l’Assemblée nationale, réclamé de longue date par les associations du secteur, comporte des avancées significatives, qui répondent en partie aux attentes. Ces associations

En effet, à la demande du Gouvernement, différents articles introduisant un soutien financier aux associations ont été retirés du texte, au motif de l’état inquiétant des finances publiques de notre pays. Pour mémoire, il s’agissait notamment de créer un fonds de garantie, d’instaurer des dispositifs d’exonération de taxes ou encore de majorer les incitations fiscales pour renforcer la générosité publique en la matière. Sans nier la réalité de notre situation budgétaire, force est de constater que la version issue des travaux de l’Assemblée nationale diminue grandement la portée du texte, mais aussi et surtout son ambition initiale.

L’autre argument avancé par le Gouvernement était le lancement d’un Beauvau de la sécurité civile, engagé en avril 2024, avec pour objectif de mener une réflexion globale sur la protection civile. Monsieur le ministre, à ce jour, et sauf erreur de ma part, seul un champ thématique parmi les cinq ouverts, autour

En ouverture de ce débat, de nombreuses questions se posent : combien de temps les bénévoles concernés devront ils encore attendre avant que cette loi ne soit votée ?

Que devons nous répondre aux sollicitations récurrentes des associations concernées dans nos départements, qui sont confrontées à des difficultés financières ou à des carences en matériel d’intervention ? Il est de notre responsabilité d’identifier les mécanismes financiers susceptibles de leur permettre de pérenniser leur organisation, mais aussi et surtout d’agir plus sereinement.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est temps d’inscrire de façon urgente l’examen de cette proposition de loi à notre agenda. J’espère que nous pourrons nous enorgueillir, à l’image de nos collègues députés, d’un vote unanime. C’est le moins que nous puissions faire pour des personnes qui agissent au quotidien pour la sécurité de nos concitoyens, de façon pleinement désintéressée, parfois au péril de leur propre vie. Il semble que le texte pourrait être inscrit à notre agenda avant l’été.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre modèle de sécurité civile, unique en Europe, repose sur une complémentarité entre professionnels, volontaires et bénévoles. Ensemble, ils assurent la protection de nos concitoyens face aux crises climatiques, sanitaires, technologiques ou géopolitiques. Avec près de 200 000 sapeurs pompiers volontaires et 200 000 bénévoles au sein des associations agréées de sécurité civile, ce modèle repose majoritairement sur l’engagement citoyen. Ces femmes et ces hommes, en parallèle de leur vie professionnelle et personnelle, choisissent de consacrer leur temps et leur énergie à la protection des autres, dans un esprit de solidarité et de dévouement qui fait la force de notre nation. La sécurité civile française est reconnue comme l’une des plus efficaces au monde. Elle repose sur un maillage territorial fort et une capacité à mobiliser rapidement des forces opérationnelles, que ce soit pour lutter contre les incendies gérer les catastrophes naturelles ou les situations de crise exceptionnelles. Pourtant, ce modèle est aujourd’hui fragilisé et confronté à de nombreux défis. Il est fondamental de garantir la pérennité du volontariat et du bénévolat en sécurité civile.

à des contraintes administratives incompatibles avec leur engagement. Si cette interprétation venait à s’imposer, elle pourrait décourager des vocations, complexifier les conditions d’engagement et affaiblir notre capacité de réponse aux crises. Notre assemblée a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce sujet. Elle a plaidé pour une directive européenne spécifique encadrant l’engagement citoyen bénévole et volontaire, afin de préserver le statut des intéressés et d’éviter leur requalification par le droit du travail. Le Gouvernement soutiendra t il une directive européenne spécifique pour protéger le volontariat de sécurité civile contre une telle requalification ? Avec Avec leurs 200 000 engagés, ces associations jouent un rôle fondamental dans le secours d’urgence, l’appui aux populations sinistrées, la formation aux gestes qui sauvent et l’encadrement des grands événements.

volontaires. Je pense notamment à la facilitation de leur disponibilité auprès des employeurs et à la bonification de trimestres pour la retraite, ainsi qu’à la valorisation de leur engagement dans la formation et dans les parcours professionnels. Mais ces dispositifs ne bénéficient pas aux bénévoles des AASC,

t il la création d’un véritable statut de bénévole de sécurité civile, garantissant une meilleure conciliation entre engagement, vie professionnelle et vie familiale ? Enfin, il est impératif d’assurer un financement stable et durable aux associations agréées de sécurité civile. Ces structures, qui sont essentielles à notre capacité de réponse aux crises, fonctionnent souvent avec des moyens précaires, reposant sur des dons, des subventions ponctuelles ou des mécénats incertains. La proposition de loi de notre collègue député Yannick Chenevard, adoptée par l’Assemblée nationale le 27 mars 2024 et en attente d’examen au Sénat, contient des avancées notables, comme la création d’un fonds de garantie assurant un financement pérenne des AASC, l’extension de certaines incitations fiscales, le bénéfice de déductions de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et l’exonération de taxe foncière

d’identifier des solutions concrètes. Quelles leçons le Gouvernement tire t il de ce travail ? Quelles mesures découleront de ces échanges et sous quels délais ? Il est de notre responsabilité de nous hisser à la hauteur des défis que notre sécurité civile, pilier

pour ne pas dire indispensable, « la protection des personnes, des animaux, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes Ces actions passent par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées. le modèle français, à la fois hybride et original, permet à plus de 250 000 sapeurs pompiers, à plus de 13 000 militaires des bataillons de marins pompiers de Marseille et sapeurs pompiers de Paris, aux 1 500 sauveteurs, pilotes d’avion et d’hélicoptère et aux 200 000 bénévoles de concourir

Mais force est de constater que notre modèle présente de sérieux signes de fatigue. Tout d’abord, cet essoufflement est dû à une pression opérationnelle exponentielle, impose des réponses adaptées et une meilleure coordination des différents acteurs de la sécurité civile. Je pense aux jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), aux interventions pour secours aux personnes, qui ne cessent de se

combien il est difficile pour eux de concilier l’engagement associatif avec les vies professionnelle et personnelle. Crise du sens pour les électeurs, crise du sens pour les salariés et, logiquement, crise du sens pour les bénévoles : le don de soi ne va plus de soi…

sur les missions à assurer, en insérant davantage encore ces bénévoles dans la chaîne de secours et de gestion des crises ; sur les recrutements, en se donnant les moyens de fidéliser les effectifs ; et sur la reconnaissance que la Nation doit à ces personnes, qui donnent de leur temps pour protéger La crise du sens est indissociable du manque de reconnaissance. C’est d’ailleurs l’objet de la proposition de loi de Yannick Chenevard, député du Var, texte adopté par

des démineurs et des personnels administratifs. Les membres des associations agréées font évidemment partie intégrante de la grande famille de la sécurité civile. Madame Schillinger,

nous permettent en effet de donner un coup de projecteur sur l’engagement de 200 000 de nos concitoyens au sein des associations agréées de sécurité civile. Ces bénévoles jouent un rôle fondamental

les bénévoles de la sécurité civile ne sont pas forcément les plus visibles. Ils jouent pourtant un rôle très important au quotidien sur notre territoire, que ce soit à l’occasion de missions d’assistance,

Chaque fois, les bénévoles de la sécurité civile ont répondu présents et répondent présents. Nous avons besoin aujourd’hui de leur engagement. Nous en aurons besoin davantage encore demain, avec l’augmentation des risques en tout genre.

Dans cette perspective, la création d’un label « employeur partenaire des associations agréées de sécurité civile » permettrait de reconnaître l’engagement des employeurs, qui doivent par ailleurs trouver une forme de compensation

Les associations de sécurité civile peinent à recruter et à fidéliser. On ne peut faire peser cette responsabilité sur des salariés isolés. Ensuite, cette proposition de loi

Parce que le territoire est complètement dépassé et non outillé, la préfecture s’organise, publie un arrêté d’interdiction et mobilise les premières forces de sécurité civile de l’État : services de la préfecture, gendarmerie, pompiers, procureur. Par ailleurs, elle réquisitionne en urgence les associations agréées de sécurité civile.

l’activité de secourisme lors d’événements publics autorisés doit être facturée auprès de l’organisateur de l’événement. À ce titre, nous devons nous demander comment mieux accompagner les associations agréées de sécurité civile,

Aujourd’hui, les recettes des formations et des prestations de service de secourisme ne permettent pas d’assurer les achats d’équipements et les investissements nécessaires aux activités des associations agréées de protection civile, en particulier celles qui font l’objet de réquisitions préfectorales.

en effet l’occasion d’évoquer, pour mieux le louer, la singularité et l’originalité du modèle de sécurité civile à la française. En effet, si la France peut s’enorgueillir de compter un corps de 255 000 sapeurs pompiers, il convient de relever que 212 000 d’entre eux sont des sapeurs pompiers volontaires et 43 000 des sapeurs pompiers des sapeurs pompiers professionnels. Ce soir, il s’agit de mettre à l’honneur ces 255 000 femmes et hommes qui s’engagent pour sauver des vies, pour lutter contre les incendies et pour faire face aux inondations. Ce débat nous donne aussi l’occasion de saluer l’engagement des centaines de milliers de bénévoles qui participent au déploiement de nos forces de sécurité civile pour porter secours et assistance à celles et ceux qui sont confrontés à un accident ou à un incendie. Je veux bien sûr parler des 200 000 bénévoles engagés dans les associations agréées de sécurité civile, des bénévoles des comités communaux feux de forêt, des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer, qui œuvrent sur nos côtes, notamment

Collaborateurs occasionnels du service public, ils sont des relais, des sentinelles, des gardiens et des acteurs à part entière de la sécurité civile

Se former, c’est monter en compétence et obtenir une meilleure reconnaissance de la part des différents acteurs institutionnels comme de la part des employeurs. L’enjeu de la montée en compétences suppose que les associations agréées de sécurité civile disposent des moyens financiers nécessaires à leur existence,

Sdis est tout aussi prégnant. Tout en préservant la distinction entre les bénévoles de sécurité civile et les sapeurs pompiers volontaires, il convient de faire partager aux uns et aux autres une culture commune, d’un point de vue tant déontologique qu’opérationnel, lors des interventions. Monsieur le ministre, ce débat me donne aussi l’occasion d’insister sur les défis auxquels notre sécurité civile à la française doit faire face. Le premier défi concerne la directive européenne sur le temps de travail. Ce texte reste une épée de Damoclès qui inquiète et trouble la sérénité des soldats du feu. quelles indications pouvez vous nous donner quant à l’adoption d’une directive spécifique visant à protéger l’engagement bénévole et volontaire dans le domaine de la protection civile ? Le deuxième défi concerne le renouvellement et la massification de nos forces de sécurité civile. Nous devons y parvenir pour faire face au vieillissement de la population, donc à l’augmentation constante des interventions pour secours à personne à domicile – à la suite d’accidents domestiques ou de chutes – ou sur la voie publique. Je rappelle que les missions de secours d’urgence aux personnes représentent 84 % des missions réalisées par les sapeurs pompiers au quotidien. À la réalité démographique liée à la pyramide des âges s’ajoute une réalité climatique, l’augmentation des inondations et des épisodes méditerranéens ou cévenols, sans parler des cyclones auxquels nos compatriotes ultramarins doivent de plus en plus faire face. Comment répondre à la crise des vocations, notamment dans le monde rural ? Comment recruter et conforter le maillage territorial pour renforcer la proximité des services de sécurité civile et garantir une réponse rapide et efficace des urgences ?

communauté d’agglomération de La Porte du Hainaut à bloquer, temporairement, un financement de quasi 8 millions d’euros. Si l’on pense bien sûr aux sapeurs pompiers, on oublie souvent, bien trop souvent, les 200 000 bénévoles des associations agréées de sécurité civile. bénévole depuis mes 16 ans dans l’une de ces associations, je ne connais que trop bien leur importance dans la capacité de résilience de la France. Nous leur devons beaucoup. Emmanuel Macron l’a d’ailleurs reconnu le 6 octobre 2017, quand il a considéré à juste titre que ces bénévoles « incarn[aient] le visage d’une France solidaire, ouverte, généreuse, d’une France qui n’a pas peur, même dans ces pires moments

Nous le savons, lorsque, en partie grâce à eux, les jeux Olympiques et Paralympiques se déroulent dans de bonnes conditions. Nous le savons encore, lorsque, dans le département du Nord, à Merville, ils sont intervenus en soutien des élus et des pompiers lors des dernières inondations.

Quelle reconnaissance pour le bénévolat de ces femmes et de ces hommes, qui ont pour seul intérêt la capacité de résilience de la France ? La proposition de loi du député Yannick Chenevard, que j’ai connu en un autre temps, avant nos engagements politiques respectifs, moi, simple bénévole à la protection civile, lui, président bénévole de la Fédération nationale de protection civile, est une réponse à ces enjeux.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne peux commencer mon propos sans rendre un hommage appuyé au plus de 250 000 bénévoles des associations agréées de sécurité civile. en effet respect et remerciements pour leur dévouement et leur engagement sans faille au service de tous. Ils forment le pilier indispensable de notre modèle de protection des populations. À tous, un grand merci ! Alors que notre territoire doit affronter de nombreux défis, nous savons que nous pouvons compter sur chacun d’entre eux. Ce sont eux qui s’engagent au quotidien afin d’accompagner, protéger, secourir, soigner ou encore réconforter les sinistrés et les blessés. Ce sont eux qui se sont mobilisés lors de la crise du covid 19 afin d’organiser et de coordonner les campagnes de dépistage et les centres de vaccination. Ce sont eux, encore, qui sont venus au secours des habitants du Nord, lorsque ce département et celui du Pas de Calais voisin ont été touchés par de violentes inondations à la fin de l’année 2023. Ce sont eux, enfin, que nous avons retrouvés cet été, à Paris, à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques, sur la grande majorité des sites qui accueillaient des épreuves. La Nation leur doit beaucoup. Ils sont indispensables à notre société. C’est pourquoi il est incontournable de réfléchir et de travailler à mieux reconnaître l’engagement des membres de cette communauté du secours, dont les associations constituent un véritable maillage, une véritable richesse. Je pense notamment à la Croix Rouge française, à la Société nationale de sauvetage en mer, à la Fédération nationale de protection civile ou à la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Je ne peux les citer toutes, mais ces associations constituent un tissu dense sur l’ensemble de notre territoire.

Comment permettre aux associations de sécurité civile de répondre avec davantage d’efficacité aux sollicitations toujours plus nombreuses des pouvoirs publics ? Comment encourager, faciliter et amplifier l’indispensable engagement de citoyens au service de notre nation ? Pour répondre au mieux à l’ensemble de ces défis, une meilleure reconnaissance du rôle de tous ces bénévoles est primordiale. Nous pourrons ainsi disposer d’un solide pilier de bénévoles mobilisables pour secourir les populations victimes ou sinistrées. Monsieur le ministre, envisagez vous de permettre à tous ces bénévoles de sécurité civile d’acquérir des droits comptabilisés en euros sur le compte personnel de formation au titre des activités de volontariat recensées au travers de l’engagement citoyen ?

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce soir, nous parlons reconnaissance du bénévolat de sécurité civile, à la demande, fort à propos, du groupe CRCE K. Plus que jamais, le bénévolat constitue l’un l’un des piliers essentiels du modèle de sécurité civile français. Il doit être protégé et encouragé. L’engagement individuel, l’abnégation, le courage face au danger et le sens du service des bénévoles et des volontaires sont remarquables. Je tiens à rendre hommage, ce soir, dans l’enceinte de la Haute Assemblée de notre République, aux bénévoles des associations de sécurité civile et à l’ensemble des sapeurs pompiers de France, volontaires, professionnels et militaires. Ils sont 250 000 bénévoles des associations agréées de sécurité civile. Pourtant, ils constituent encore un maillon souvent méconnu, bien qu’essentiel, de la chaîne de sécurité civile, s’inscrivant dans la continuité logique des personnels professionnels et volontaires des sapeurs pompiers, constituent les 250 000 autres Français à composer la grande famille de la sécurité civile de notre pays. Alliant bénévolat et spécialisation, les associations agréées de sécurité civile contribuent à faire vivre la culture du risque parmi la population et à augmenter sa résilience. Elles peuvent, dans certains cas, venir en appui des sapeurs pompiers

du statut créé par la loi du 3 juillet 2020. La FNSPF appelle aussi, justement, à mieux valoriser les anciens sapeurs pompiers en les incitant à rejoindre les réserves citoyennes des Sdis et en appelant à systématiser la création de réserves communales de sécurité civile dans les communes dotées d’un plan communal ou intercommunal de sauvegarde et à parfaire la connaissance des ressources bénévoles par l’autorité préfectorale. Assurer une meilleure reconnaissance des associations agréées de sécurité civile a été l’un des aspects majeurs de la proposition de loi

La Chambre haute pourrait s’enorgueillir d’inscrire rapidement à son ordre du jour cette proposition de loi qui vise à pérenniser et amplifier le bénévolat dans la sécurité civile en donnant aux quelque 600 associations agréées les moyens d’agir. Ce texte prévoit notamment de faciliter les possibilités d’absence professionnelle, entre autres, grâce à un label à destination des employeurs, et développe les pistes d’une meilleure reconnaissance de l’engagement bénévole. Comment améliorer la reconnaissance du bénévolat de sécurité civile ? Cette question, nous nous la sommes aussi posée, au sein du groupe de travail interne au groupe Les Républicains du Sénat relatif à la sécurité civile, que j’ai eu l’honneur d’animer durant dix huit mois. Dans ce cadre, nous avons souhaité mettre en avant plusieurs préconisations de bon sens. Il nous a semblé qu’il existait un retard dans la délivrance des décorations et autres marques de reconnaissance. Celui ci a commencé à être comblé durant les dernières années, d’abord au travers de la création de la médaille de la sécurité intérieure, puis par la création, dans la loi Matras de 2021, de la mention « Mort pour le service de la République ». Malgré cela, beaucoup reste encore à faire. Avec le groupe de travail, nous avons considéré qu’il serait opportun de renforcer les efforts de reconnaissance honorifique et symbolique, tant des sapeurs pompiers que des membres d’associations agréées de sécurité civile, en réfléchissant à la mise en place de critères d’attribution et en s’inspirant de l’exemple des pratiques au sein des unités militaires exerçant des fonctions de sapeurs pompiers à Paris et Marseille. Au travers de nos auditions, il nous est également apparu qu’il fallait conforter les associations de sécurité civile dans leur rôle d’auxiliaires indispensables de l’action des pouvoirs publics. Pour ce faire, notre rapport préconise aussi d’améliorer la visibilité, une meilleure communication publique, des formations aux premiers secours, de renforcer les efforts de formation des élèves du secondaire, d’associer plus étroitement les associations agréées

Toutes ces pistes, et tant d’autres, sont autant de propositions simples et de bon sens que je souhaitais apporter à notre débat de ce soir, tant le bénévolat de sécurité civile est essentiel en tant qu’organe participant grandement à la capacité de résilience de notre pays. La parole est à M. le ministre.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues,

ou encore la proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale le 25 avril 2023 par notre collègue député Chenevard, que je salue à mon tour, visent à apporter des réponses à cette volonté de valorisation et de renouvellement du volontariat.

L’extension aux bénévoles de sécurité civile des droits dont bénéficient les sapeurs pompiers volontaires depuis la loi Matras de 2021 ne doit pas créer une telle concurrence, sous peine de nuire à notre modèle de sécurité civile dans son ensemble. L’alchimie est ici essentielle

Un décret récent vise justement à simplifier les modalités d’habilitation et à alléger la charge administrative d’instruction des demandes par les préfectures, pour leur permettre de se concentrer sur leur mission de contrôle des entités habilitées et pour rendre plus lisible la réglementation

78 % des effectifs de sapeurs pompiers. Ceux ci interviennent au quotidien et au cœur des crises pour porter un secours immédiat. Les sapeurs pompiers assurent 75 % des opérations de secours, ce qui en fait le premier service d’urgence de proximité de notre pays. À leurs côtés, les associations de sécurité civile comptent environ 200 000 membres. Elles assurent des missions complémentaires de prévention, sécurisent les grands rassemblements de personnes et sont essentielles pour anticiper les crises et assurer le retour à la normale.

solution pour nos concitoyens, le dernier service public de proximité. La Cour des comptes écrivait déjà, dans un rapport de 2019, que les sapeurs pompiers compensaient la désertification médicale, en particulier dans les territoires ruraux.

monsieur le ministre,

Carrère Gée. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il est des vies consacrées à des causes plus grandes que soi, des actions qui cimentent la résilience de notre nation. L’engagement des bénévoles de la sécurité civile en est une illustration incontestable. Ils sont 250 000 femmes et hommes à répondre présents quand l’urgence l’impose pour protéger, secourir, préserver. inondations, crises sanitaires : à chaque épreuve, ils sont là. Dans les épreuves de la vie, aussi : pour avoir participé à des maraudes de la protection civile, à Paris, auprès de personnes à la rue, je sais toute leur expertise pour écouter et prendre en charge les blessures physiques comme psychiques des plus plus vulnérables. Ces bénévoles, nous en aurons toujours plus besoin et en plus grand nombre. Comme l’avait fait peu de temps auparavant l’ouragan Irma à Saint Martin, le cyclone Chido à Mayotte nous a interpellés sur la dramatique insuffisance en matière de culture du risque chez de nombreux citoyens et sur toutes les difficultés à entrer en contact avec les populations les plus vulnérables – je parle de vulnérabilité non seulement géographique, mais aussi sociale ou culturelle. Mieux reconnaître et faciliter l’engagement des bénévoles des associations agréées de la sécurité civile, faire confiance à leur expertise de terrain et à leur proximité avec la population, c’est se donner les moyens de faire vivre une solidarité en action.

faudra de nouveau évoquer des dispositions qui n’ont pas été adoptées à l’Assemblée nationale, comme le renforcement du modèle économique des associations agréées de sécurité civile ou une meilleure défiscalisation des dons. Le Beauvau de la sécurité civile, vous l’avez dit, monsieur le ministre, doit reprendre ce débat crucial et un projet de loi doit nous être présenté rapidement. Nous serons très exigeants pour nous montrer à la hauteur de l’engagement et des compétences de nos bénévoles. Monsieur le ministre, à l’heure de la multiplication et de l’aggravation des risques, je compte aussi sur le Beauvau de la sécurité civile pour accomplir des progrès décisifs en matière d’implication citoyenne.

Il est absolument incroyable que les rares outils technologiques qui ont été mis en place ne soient destinés qu’à l’information de la population, de manière totalement verticale. Pourquoi ne sont ils pas déployés pour permettre à chaque citoyen d’être acteur du secours à la Nous connaissons tous l’application « SAUV Life », qui permet à tous ceux qui sont inscrits d’être alertés si quelqu’un fait un arrêt cardiaque à proximité. Pourquoi n’a t on pas encore sur nos smartphones une application qui nous permette, par exemple en cas de catastrophe naturelle, de nous former et d’intervenir utilement dans l’attente des secours, éventuellement en étant guidés N’ayons pas peur de faire de chaque citoyen un acteur. À condition d’avoir les bons outils et les bonnes méthodes, la participation de tous conduit non pas à désorganiser la sécurité civile, mais à en démultiplier la puissance.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, étant la dernière intervenante dans ce débat et beaucoup de choses ayant déjà été dites, je ne reviendrai pas sur le contexte, les enjeux et les défis qui nous imposent aujourd’hui de mettre en place de nouvelles évolutions de notre modèle de sécurité civile et de mieux reconnaître le bénévolat de ceux qui s’y engagent. Nous sommes tous d’accord sur le fait que la pression opérationnelle ne va que s’accentuer du fait de la multiplication des crises, comme les aléas climatiques de plus en plus hors norme ou les besoins croissants de secours à la personne du fait du vieillissement de la population. Une proposition de loi a été adoptée à l’Assemblée nationale. J’espère qu’elle sera prochainement discutée dans cet hémicycle, à moins que le Gouvernement ne dépose un projet de loi plus large et plus complet encore, issu des travaux du Beauvau de la sécurité civile. La proposition de loi de notre collègue Yannick Chenevard est déjà très complète. Pour ma part, forte de ce que je connais dans le Haut Rhin, où le tissu associatif est particulièrement dynamique, je peux affirmer que, même si celui ci repose sur un engagement désintéressé, sa reconnaissance est néanmoins un pour maintenir la motivation et éviter l’épuisement des femmes et des hommes qui y consacrent leur temps. L’amélioration du statut juridique, le renforcement des formations, la bonification de la retraite, la création de droits spécifiques ou encore la mise en place d’indemnités, à l’instar de ce qui existe déjà pour les sapeurs pompiers volontaires une autre forme d’engagement que je connais bien puisqu’il y en a plus de 4 000 dans mon seul département du Haut Rhin – sont indispensables. La reconnaissance peut aussi être honorifique pour ces bénévoles, dont l’engagement repose sur un équilibre entre compétences techniques et qualités morales, garantissant un secours efficace et respectueux des personnes aidées. Comme pour nos forces de l’ordre, décerner une décoration est une façon de reconnaître de manière officielle, publique et significative leur action et leur engagement.

Concernant la promotion du 1 janvier 2024, seuls trois récipiendaires sur 2 400 l’ont reçue avec l’agrafe « sécurité civile » ou « engagement citoyen ». Au vu des dizaines de milliers de membres actifs engagés dans les 600 associations agréées de sécurité civile dans notre pays, c’est très peu, pour ne pas dire insignifiant. À titre d’exemple, dans mon département, le président de la Croix Rouge de la section des Trois Frontières est un bénévole actif depuis quarante sept ans, soit presque autant qu’une vie de travail. Un engagement d’une telle durée ne mériterait il pas d’être publiquement reconnu ? Paolo Coelho a écrit que les choses simples sont les plus extraordinaires. Je crois, monsieur le ministre, tout comme ma collègue Françoise Dumont – et comme vous l’avez vous même dit

Ces bénévoles, engagés sans attente de contrepartie financière – ma collègue Mireille Jouve a parlé tout à l’heure de « don de soi » –, se mobilisent lors de catastrophes naturelles, d’accidents majeurs ou de crises sanitaires, apportant un soutien professionnel précieux aux services de secours et aux autorités. Leur dévouement illustre une solidarité sans faille et contribue directement à la résilience de notre société face aux aléas.

Tout au long de ce débat, nous avons exploré différentes facettes de la reconnaissance du bénévolat de sécurité civile. Certains pourraient considérer que, dans la mesure où le bénévolat repose sur le principe même du désintéressement, une reconnaissance trop institutionnelle risquerait d’altérer cet esprit de volontariat. Je n’y crois pas. Je plaide plutôt en faveur d’une valorisation plus explicite de tels engagements, soulignant les compétences acquises sur le terrain, la disponibilité exigée et les responsabilités assumées, qui mériteraient une meilleure prise en compte sur le plan tant individuel que sociétal crois, d’une question de société. La reconnaissance du bénévolat peut se décliner sous plusieurs formes : une meilleure intégration des bénévoles dans les dispositifs de ce cadre civil ; un renforcement de leur formation et des moyens mis à leur distribution ; une valorisation officielle de leurs compétences dans le cadre académique ou professionnel. Il s’agit ici non pas de remettre en question le caractère altruiste de leur engagement, mais bien de reconnaître leur rôle clé dans la gestion des crises et de s’assurer qu’ils disposent des outils nécessaires pour agir.

la mise en place de dispositifs intégrant des droits à la retraite ou l’obtention de distinctions honorifiques. J’ai demandé au préfet du Pas de Calais d’honorer mes bénévoles ; si vous étiez disponible, monsieur le ministre, ce serait avec beaucoup de plaisir que je vous accueillerais à Arras. telles mesures visent non pas à transformer le bénévolat en un travail rémunéré, mais à le valoriser et à encourager un engagement pérenne. La reconnaissance du bénévolat de sécurité civile doit s’inscrire dans une réflexion plus large sur le rôle des citoyens dans la gestion de crise. Dans un monde où les crises sont de plus en plus fréquentes et complexes, je pense qu’il est essentiel d’encourager la participation active de tous à la sécurité collective ; nous parlons presque de citoyenneté.

la nécessité de mieux reconnaître l’apport essentiel des bénévoles de la sécurité civile. Il appartient désormais aux décideurs, aux organisations et même aux citoyens de transformer ces réflexions en actions concrètes pour que cet engagement soit non seulement reconnu, mais aussi renforcé, dans l’intérêt de tous. Notre débat illustre à quel point le bénévolat est une force indispensable en période de crise venant compléter et renforcer l’action de services publics.

Merci,